Monsieur le président,

qui travaillent pour assurer la sécurité de tous au péril de leur vie. S'agissant des éléments financiers, la mission « Anciens combattants, mémoire et liens

900 millions d'euros ; pour 2021, les crédits demandés baissent de 70 millions environ. Au total, les crédits des trois

la commission des affaires sociales s'est, comme chaque année, saisie pour avis des crédits de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », qui correspondent essentiellement à des prestations sociales de reconnaissance ou de réparation. Comme chaque année, la baisse du nombre de bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité ou de la retraite du combattant, qui sont, pour leur grande majorité, des anciens de la guerre d'Algérie ou des conflits antérieurs, entraîne une réduction des dépenses correspondantes. En effet, le nombre de cartes du combattant attribuées au titre des opérations extérieures est chaque année dix fois moins important que le nombre d'anciens combattants qui décèdent. Cette baisse régulière des dépenses de guichet en faveur des anciens combattants permet au Gouvernement de donner satisfaction à certaines des demandes, parfois anciennes et récurrentes, du monde combattant. Ainsi, en 2021, le niveau d'invalidité ouvrant droit à une majoration de la pension de réversion sera abaissé. Cette mesure devrait bénéficier à moins de deux cents personnes et coûter 1 million d'euros. Il me semble qu'un chantier plus structurel mérite d'être ouvert, s'agissant des modalités d'indexation du point de PMI, qui détermine le montant de l'ensemble des prestations servies aux anciens combattants. Je sais, madame la ministre, que vous avez annoncé la création d'un groupe de travail associant des parlementaires et qui devrait se réunir prochainement. D'autres demandes existent en matière de politique de mémoire et de reconnaissance. Alors que certaines d'entre elles seront abordées à l'occasion de la discussion des amendements, des avancées sont également attendues par ceux qui sont déployés en opération intérieure- Sentinelle ou Harpie, par exemple -, comme les réservistes, afin que le titre de reconnaissance de la Nation leur soit attribué. S'agissant de la politique de mémoire, je note que ces dépenses, qui avaient été financées en 2020 par un prélèvement sur la trésorerie de l'ONAC-VG, sont réintégrées dans le budget de l'État. Nous n'en doutions pas, mais je salue, madame la ministre, le respect de l'engagement pris par le Gouvernement sur ce point. Par ailleurs, la population des anciens combattants sera, dans les années à venir, plus jeune et composée d'anciens soldats de métier, dont les attentes ne seront pas les mêmes que celles des anciens appelés de la guerre d'Algérie. La politique en leur faveur devra évoluer et pourrait nous conduire à nous interroger sur la notion même d'ancien combattant, à laquelle il faudrait peut-être préférer celle, plus large, de « monde combattant », voire de « combattant Les crédits dédiés aux liens armées-jeunesse tiennent compte du report sur 2021 d'une partie des Journées défense et citoyenneté qui n'ont pu être organisées en 2020 en raison de la situation ; ils tiennent également compte de l'augmentation de la cible des engagements en service militaire volontaire. J'en profite pour attirer l'attention du Gouvernement sur ces dispositifs, qui doivent permettre de mieux déceler les situations de fragilité chez les jeunes et, en particulier, d'identifier les jeunes aidants et de leur apporter le soutien nécessaire. Pour conclure, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission, ainsi que de l'article 54. Mes chers

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis le mois de mars, notre pays traverse une épreuve, durant laquelle il a été beaucoup question de première ligne, de privation de liberté et- hélas ! -de deuil. Mieux que quiconque, les anciens combattants savent ce qu'est le sacrifice. Ils savent aussi que, au bout du tunnel, il y a l'espoir du retour à une vie normale et que, par-delà les drames, restera le souvenir des moments de fraternité. Je pense en particulier aux élans de solidarité exprimés par des applaudissements, au plus fort de la crise, en direction de nos personnels soignants partis au combat contre un ennemi invisible, un virus ; certains d'entre eux avaient peur d'être infectés, mais ont néanmoins servi leur noble vocation. Les hommages, quelle que soit leur forme, sont fondamentaux, car ils nous rappellent combien l'addition des courages individuels peut déterminer le destin de tout un pays. Daniel Cordier l'avait bien compris, en risquant son propre destin au service de la liberté de tous les Français. Ce résistant de la première heure vient de nous quitter, à tout juste cent ans, en digne représentant du « peuple de la nuit », aurait dit André Malraux. L'hommage qui lui a été rendu le 26 novembre dernier succède à l'entrée au Panthéon de « ceux de 14 »

le devoir de mémoire est plus que jamais nécessaire face à la disparition des grands témoins des conflits du XX siècle. Je partage aussi leur idée d'associer davantage à cette politique l'engagement des militaires en OPEX, qui est de plus en plus difficile, en particulier au Sahel.

Je souhaite saluer la mesure nouvelle intéressant le droit à réparation : l'article 54 du projet de loi de finances prévoit une majoration de la pension du conjoint survivant d'un titulaire d'une pension militaire d'invalidité, dont l'indice était au moins égal à 6 000 points.

Il serait en effet souhaitable de trouver un mode d'indexation qui préserve les droits des anciens combattants. Nous le leur devons, car, comme le Président de la République l'a rappelé le 11 novembre dernier, « leur sacrifice dit notre dette et nos devoirs ». En attendant, le groupe RDSE votera les crédits de cette mission. La

très satisfait. Un ministère en tant que tel demeurera utile tant que les contentieux ne seront pas totalement réglés. Il convient d'ailleurs qu'il en soit ainsi, s'agissant des réparations pour services rendus à la République. Depuis des années, nous oeuvrons pour que le monde combattant obtienne réparation ; je veux rappeler que cette année verra la mise en oeuvre de la mesure tant attendue de l'extension de la demi-part fiscale en faveur des conjoints survivants âgés de 74 ans et plus, dont le conjoint percevait la retraite du combattant. La principale mesure annoncée concerne l'extension du nombre de veuves de grands invalides de guerre qui pourront bénéficier d'une augmentation de leur pension. C'est une bonne chose.

Il demeure toujours des inégalités et je déplore une nouvelle fois l'attitude du Gouvernement qui semble jouer la montre en ce qui concerne la troisième génération du feu- ce sont les derniers à avoir servi dans le cadre de la conscription

Madame la ministre, le coût des améliorations à apporter dans le cadre de l'égalité des droits entre acteurs d'un même conflit ou entre générations du feu ne bouleverserait pas sensiblement l'équilibre du budget de notre pays. Faire des économies de bouts de chandelle n'est pas tolérable envers des militaires qui ont servi leur patrie au péril de leur vie, de leur santé, de leur vie de famille, de leur vie professionnelle et qui n'avaient pas d'autre choix que de servir, en répondant à l'appel pour combattre Avec un taux de mortalité qui ne peut que s'accroître et qui est certainement voisin de 6 % pour la troisième génération du feu, une baisse du budget total de 3,4 pourrait être considérée comme acceptable. Hélas, tout en relevant les points positifs de la réparation, nous ne pouvons pas nous en satisfaire. En effet, des mesures en trompe-l'oeil, comme des transferts de budget,

L'inscrire dans ce PLF réglerait totalement ce point de contentieux. Nous sommes toujours dans l'attente de la constitution d'une commission tripartite chargée de trouver une solution au dérapage entre l'évolution des prix à la consommation, hors tabac, et celle de la valeur du point de PMI. Il s'agit d'une urgence absolue, tant cette différence porte atteinte, notamment, aux titulaires de PMI dont le handicap n'est pas compensé à sa juste valeur.

En effet, l'ensemble des politiques publiques qui contribuent à pérenniser les liens entre la Nation et le monde combattant est décliné au sein de cette mission, à travers trois programmes budgétaires, dont les principales orientations ont été évoquées par mes collègues.

La trajectoire des crédits de paiement prévus pour 2021 confirme la baisse structurelle et naturelle de la population concernée par les pensions militaires d'invalidité et par la retraite du combattant, qui sont les deux dispositifs budgétaires les plus importants de la mission.

des attentats terroristes qui frappent la République. Il est également fondamental que l'ONAC-VG renforce ses missions afin de valoriser davantage les combattants de la quatrième génération du feu et de toutes les opérations extérieures ; il doit aussi mettre en place une action particulière pour les dissidents ultramarins. Les économies réalisées devraient servir, même partiellement, à renforcer les actions en faveur du monde combattant. Je déplore que cela ne soit pas le cas.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'examen des crédits de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » constitue toujours un moment particulier, car derrière les chiffres et les colonnes, les programmes et les lignes de ce budget, se concentrent les vies de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui consentent pour notre pays au sacrifice suprême. Cette mission finance les actions de reconnaissance en faveur du monde combattant, les politiques de renforcement du lien entre l'armée et la Nation et l'indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette année encore, les crédits de la mission sont en diminution d'environ 3 % et sont désormais inférieurs à 2,1 milliards d'euros. Toutefois, cette chute est pour partie la conséquence de la diminution du nombre de bénéficiaires de la retraite du combattant et de la pension militaire d'invalidité. Pour 2021, plus encore qu'auparavant, les attentes des anciens combattants et de leurs familles sont fortes et légitimes la mesure de revalorisation prévue cette année consiste en l'abaissement du seuil d'invalidité nécessaire à l'obtention de la majoration de la pension de réversion du conjoint survivant d'un grand invalide de guerre. Cette mesure était attendue. Ainsi, une veuve de grand invalide de guerre pourra bénéficier d'un supplément de pension militaire d'invalidité : si son conjoint décédé avait bénéficié, sur cette pension, de 6 000 points, ce nombre passera à 10 000. Je tiens aussi à saluer d'autres avancées en ce qui concerne la jeunesse, notamment la hausse satisfaisante de la cible d'incorporation du service militaire volontaire. dispositif d'insertion très performant accueillera 1 200 jeunes en 2021, soit 200 de plus qu'en 2020, grâce à une évolution de son organisation. Pour l'année 2022, l'objectif est d'accueillir 1 500 jeunes. Par ailleurs, les crédits dévolus à la politique de mémoire augmentent nettement. Cette hausse bénéficie principalement à l'aménagement et à la rénovation des sépultures de guerre et des hauts lieux de la mémoire nationale en France, en Algérie et au Maroc. Je ne peux que me féliciter de cet effort important qui permettra de conserver ces lieux de transmission dans un état décent. Avant de conclure, je voudrais exprimer toute ma gratitude aux anciens combattants qui ont été très durement éprouvés par la crise sanitaire. Ceux qui font vivre le monde combattant sont souvent des personnes d'un certain âge et l'annulation prolongée des cérémonies et des manifestations commémoratives a mis un coup d'arrêt brutal à leur travail de transmission, les privant également de rencontres particulièrement essentielles pour leur vie sociale. Madame la ministre, mes chers collègues, si ce budget diminue de 70 millions d'euros, il demeure néanmoins satisfaisant. Les droits en faveur des anciens combattants et de leurs ayants droit sont maintenus, voire étendus dans certains cas- je m'en réjouis. Il nous faudra toutefois demeurer particulièrement vigilants quant aux travaux de la commission tripartite- État, Parlement, associations -prévue au dernier trimestre 2020 qui doit examiner l'évolution du point de pension militaire d'invalidité que nous appelons de nos voeux. Le groupe Les Indépendants-République et Territoires votera les crédits de cette mission.

la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » voit ses crédits baisser, comme chaque année. Cela s'explique par la diminution du nombre de bénéficiaires, mais pas uniquement. En tout cas, certaines personnes attendent toujours de bénéficier de ces crédits. Je pense notamment à la reconnaissance de certains harkis supplétifs de statut civil de droit commun attendent toujours une aide de seulement 4 150 euros. Cette problématique se pose chaque année. À l'Assemblée nationale, nos collègues députés ont déposé des amendements pour corriger cette injustice ; on leur a opposé tout un tas d'arguments contestables

extension, la jurisprudence du Conseil d'État relative à la désignation explicite ou implicite des bénéficiaires d'une mesure adoptée par le Parlement est en leur faveur et ni le Conseil d'État ni la CEDH n'a rendu de tels jugements.

Ce n'est pas la seule injustice, sur laquelle je souhaite revenir. L'an dernier, le Parlement a adopté une disposition, qui prendra effet au 1 janvier prochain, élargissant aux veuves de 74 ans et plus le bénéfice d'une demi-part fiscale supplémentaire, à la condition que leur mari, que leur mari, titulaire de la carte du combattant ou d'une retraite du combattant, soit décédé à partir de 65 ans. Mais des femmes, dont le mari est parti avant 65 ans ? Cet effet de seuil crée une rupture d'égalité déplacée ; une telle situation requiert non pas des mesures ciblées, comme vous le répétez, mais une mesure globale d'équité. Après les anciens combattants, je souhaite aborder le lien entre le monde combattant et la Nation.

les jeunes Français doivent, en trois heures trente seulement, découvrir les enjeux qui mènent la France à développer un appareil de défense et les caractéristiques de celui-ci, passer des tests de langue française pour repérer les jeunes qui auraient besoin d'être accompagnés, apprendre les gestes de premiers secours et suivre une formation élémentaire de sécurité routière

Alors que les derniers poilus se sont éteints, que Daniel Cordier vient de nous quitter et qu'il ne reste plus qu'un Compagnon de la Libération, la question de la transmission de la mémoire des guerres mondiales et, plus largement, de la mémoire du XX siècle devient de plus en plus prégnante. ce titre, je salue la mission confiée à Benjamin Stora sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Suivant cet exemple, je crois qu'il est temps d'engager le pays dans une réflexion beaucoup plus large sur sa politique mémorielle. L'État ne remplacera jamais la transmission qui pouvait s'opérer, dans les familles, par les témoins directs du siècle passé néanmoins, il faut imaginer des moyens pour améliorer la transmission mémorielle auprès des jeunes générations. J'en profite pour saluer le travail important des associations de souvenir.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « en fait de souvenirs nationaux, les deuils valent mieux que les triomphes, car ils imposent des devoirs, ils commandent l'effort en commun. Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore », disait Ernest Renan en 1882. Le devoir de mémoire est donc au centre de ce qui nous permet de faire Nation.

Néanmoins, cette année encore, cette baisse est essentiellement le reflet de la diminution naturelle du nombre de bénéficiaires des pensions militaires d'invalidité et de la retraite du combattant. Cela dit, cette mission ne concerne pas que les anciens combattants elle intègre aussi les victimes indirectes des grands drames nationaux. Le programme 158, « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale », aide à la résilience des victimes de spoliations antisémites et soutient les orphelins. Notre objectif est désormais d'améliorer le délai de paiement des dossiers validés. Les crédits de ce programme s'établissent à 93 millions d'euros, dont un peu moins de 2 millions d'euros de dépenses de fonctionnement. La crise sanitaire a bien sûr eu un impact énorme sur le déroulement des programmes de la mission. Tout d'abord, cette pandémie a différé à 2021 et 2022 les chantiers sur les sépultures de guerre, partout sur le territoire national. De plus, alors que des cérémonies majeures ont été affectées en 2020, le même schéma risque de se produire en 2021. Ainsi, les crédits dédiés aux commémorations s'élèvent, comme en 2020, à 4 millions d'euros.

d'orientation sont maintenus- nous nous en félicitons. En effet, cette journée assure la diffusion de l'esprit de défense auprès des jeunes Français ; elle est essentielle à la cohésion nationale. Le PLF pour 2021 renforce également les crédits du programme 167, avec la réalisation d'une JDC en ligne et d'une journée Défense et mémoire nationales dans le cadre du service national universel. Expérimentée en 2019 et en 2020,

retrace la majoration de 360 points de la pension de réversion aux conjoints survivants, dont les bénéficiaires seront plus nombreux. Ce programme intègre également l'extension de l'attribution de la carte du combattant aux forces françaises présentes en Algérie entre 1962 et 1964, dite carte « 62-64 ». Enfin, il s'attache à la modernisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) et de l'Institution nationale des Invalides, avec la dématérialisation de l'ensemble des démarches spécifiques au monde combattant. Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera en faveur de ces crédits. Par ailleurs, plusieurs associations attendent la création d'une agrafe pour la médaille de la défense nationale. agrafe serait accessible au personnel civil ou militaire ayant participé aux essais nucléaires entre 1960 et 1996 sur les sites du Sahara et de la Polynésie française. Madame la ministre, pouvez-vous nous assurer que la réalisation de ce projet est toujours d'actualité ? La parole

un honneur, parce que tous les maires ont le coeur qui bat un peu fort, lorsqu'ils se tiennent devant le monument aux morts de leur commune. Les anciens combattants, la mémoire, les liens avec la Nation font partie de leur ADN. un honneur que de porter les intérêts des combattants d'hier et des anciens combattants de demain. « Je hais la guerre, mais j'aime ceux qui l'ont faite », écrivit Dorgelès. Dans le cadre des réunions préparatoires, j'ai participé à plusieurs auditions qui m'ont permis de mesurer l'importance et le poids des associations. Il y eut des temps forts. J'ai noté cette phrase, qui m'a vivement atteinte : « C'est dégradant de toujours réclamer la justice pour nos camarades. » Madame la ministre, je ne souhaite pas que vous preniez cette flèche pour vous, car je sais votre dévouement, votre sincérité et votre disponibilité au service du monde combattant.

Les crédits dédiés à la mémoire progresseront de plus de 6 millions d'euros, retrouvant ainsi un niveau proche de celui des années antérieures. Je suis très sensible également à la progression de 3,5 millions d'euros des crédits destinés à l'entretien des sépultures de guerre et des hauts lieux de mémoire nationale. La restauration des sépultures, y compris dans nos cimetières ruraux, représente un travail colossal. Le recensement, le conventionnement avec les maires et la mise en oeuvre, puis la réalisation des travaux, voilà une entreprise jamais achevée, qui demande une énergie folle, mais qui est hautement symbolique. J'attire votre attention, madame la ministre, sur le fait que, si le monde associatif est dans les territoires le bras armé de la mémoire, il doit être fortement soutenu. Quant aux crédits

» de la mission, le programme 169, présente une trajectoire budgétaire probablement unique, que je trouve personnellement assez troublante. Tablant sur ce que le comptable appelle pudiquement une « baisse naturelle », on accorde au monde combattant, au fil de l'eau et des décès, une enveloppe qui va diminuant. Il arrive que des demandes, parfois très anciennes, mais toujours légitimes- des « marronniers » -, finissent par être satisfaites au détour de cette évolution arithmétique favorable au budget de l'État. La reconnaissance nationale ne consisterait-elle pas plutôt en l'analyse de ce que l'on doit objectivement à ces hommes et à ces femmes ? Inverser la réflexion, partir du chiffrage des droits, au lieu de donner des ristournes sur les sommes qui se libèrent, voilà qui éviterait cette négociation annuelle effectivement dégradante- il faut le reconnaître -, qui ramène les associations devant le législateur pour une forme de marchandage ; ce ne sont pourtant pas des négociations syndicales Les hécatombes humaines de la Grande Guerre ont fait prendre conscience à l'État du besoin de reconnaissance de la population vis-à-vis des victimes. Le droit à reconnaissance et à réparation est devenu la règle pour tous les soldats meurtris dans leur chair au cours de leurs missions au service de la Nation, pour les civils, victimes collatérales de la guerre ou du terrorisme, mais aussi pour les orphelins et les veuves. C'est une règle imprescriptible. Alors, par respect pour ce principe, le budget du monde combattant pourrait avoir une forme de stabilité, qui serait cohérente. Au lieu d'être une variable d'ajustement, il pourrait intégrer, par exemple, l'ajustement automatique du point de pension, qui accuse toujours un retard chronique ; c'est une grave injustice. On ne peut pas faire aux anciens combattants de vibrants discours d'hommage, sans corriger ces distorsions. ces distorsions. Comme le demandent les associations, il faut étendre le droit à reconnaissance aux ascendants, au même titre qu'aux descendants. Alors que des avancées significatives ont déjà eu lieu grâce à vous, il subsiste des incohérences, que l'évolution budgétaire de cette mission aurait dû permettre de compenser. À ce jour, les veuves de titulaire d'une carte d'ancien combattant sont toujours exclues du bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire, si leur époux est décédé avant de percevoir la retraite d'ancien combattant. Sont également exclues, quel que soit l'âge de décès de leur époux, celles qui ont moins de 74 ans. Pourquoi ? Madame la ministre, ne nous arrêtons pas au milieu du gué ! Le monde combattant évolue. On ne peut gérer ce dossier comme étant en voie d'extinction. Les opérations extérieures amèneront des besoins nouveaux, des situations nouvelles ; il faut sanctuariser ce budget, arrêter son érosion, qui n'est pas une fatalité. Quel est l'avenir du droit à reconnaissance et à réparation ? Il se traduit, actuellement, par un certain nombre modalités fiscales, qui doivent simplement être justes, compréhensibles, cohérentes, sans effet de seuil et pérennes. La reconnaissance, c'est aussi une pension ajustée, stable, non négociable. Quel est l'avenir du budget des anciens combattants ? Devenir, au fil du temps et des décès, un « ancien budget », éteint ou presque, en même temps que les anciens d'Algérie ? Changeons son intitulé qu'il cesse d'être le budget des anciens quelque chose et devienne simplement le budget de la reconnaissance nationale, si cela permet d'enrayer cette morbide décrue. « L'homme est une machine à oublier », a écrit Maurice Genevoix

Merci Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avant de commencer, je tiens à rendre un hommage appuyé à tous les anciens combattants et aux membres des associations patriotiques, dont nous connaissons le travail, l'engagement et les valeurs, valeurs, d'autant que, cette année, l'organisation des commémorations a été totalement bouleversée. D'ailleurs, la façon de commémorer en temps de pandémie est une réflexion qui doit être menée. Une Nation qui rencontre de graves crises a besoin de se retrouver et de souder sa jeunesse au travers d'une mémoire qui puisse être source d'espoir et de courage. Madame la ministre, nous saluons les efforts réalisés pour moderniser et adapter les outils de communication et les supports permettant une meilleure transmission et une plus grande accessibilité de notre patrimoine mémoriel. Le volet numérique est un levier très utile pour développer le lien armées-Nation ; il représente une vaste ressource pour le monde enseignant et éducatif, pour qui la tâche est difficile face aux communautaristes qui refusent toute appartenance à la Nation et face à ceux pour qui mémoire rime avec repentance et, finalement, avec ignorance. Toutefois, le numérique ne doit être qu'un outil, un complément ; il ne peut se substituer à la force de la réunion et de la rencontre des citoyens, lors des commémorations et des formations censées forger l'esprit de défense et développer la citoyenneté. Cela m'amène naturellement à l'organisation de la Journée défense et citoyenneté. Le déploiement d'un dispositif en ligne pose question : va-t-il se substituer définitivement à l'organisation d'une journée en présentiel ? C'est une question importante, car le brassage entre jeunes issus de différents milieux sociaux et culturels partie de la citoyenneté. Nous observons bel et bien un rétrécissement des ambitions de cette journée, dont la pertinence tend à disparaître dans le format à venir. Que penser de cette numérisation, alors que nous entrons dans la deuxième année d'expérimentation

Si le SNU était une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron, en 2017, un tel dispositif, s'accompagnant d'un doublement des crédits en 2021, ne peut s'affranchir d'un véritable débat ni d'un vote de la représentation nationale. de la mission « Sport, jeunesse et vie associative », mais il est difficilement compréhensible que son périmètre et son pilotage soient autant dissociés de votre ministère. J'en viens maintenant aux crédits en eux-mêmes. Nous assistons, cette année encore, à la baisse de la dotation, de 3,2 %, attribuable dans sa quasi-totalité au programme 169, « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant La baisse démographique explique cette évolution, mais ne saurait justifier cette tendance qui est baissière depuis 2012. Elle devrait au contraire servir à aider davantage les anciens combattants et à renforcer les actions de sensibilisation auprès des jeunes, dont le lien avec la mémoire tend à s'estomper lorsqu'ils quittent l'école. Au nom du groupe Les Républicains, je regrette que les anciens combattants n'aient pas été reconnus à leur juste valeur. Je pense bien sûr à la revalorisation de la retraite du combattant et à l'augmentation du point de la

presque parler d'aumône ! Ce soutien est d'autant plus nécessaire que la paupérisation des anciens combattants retraités s'est accrue en 2020 avec la crise sanitaire, alors que leurs sources de revenus sont déjà très limitées. Avant de conclure, je veux revenir sur l'ONAC-VG et sur le contrat d'objectifs et de performance 2020-2025. Cet office doit pouvoir poursuivre sa mission avec les moyens adaptés et au plus près de ses bénéficiaires. Son ancrage territorial et départemental ne saurait être remis en cause. De même, le service et l'accompagnement des anciens combattants doivent rester des points majeurs de son action. Nous resterons donc vigilants sur la rénovation annoncée

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j'interviens sur cette mission budgétaire, parce qu'elle est essentielle à mes yeux. Fille et petite-fille d'instituteurs, j'ai toujours participé aux commémorations, avec les enfants de ma classe. C'était l'usage, à l'époque, et c'était bien, parce que nous étions très émus au son de. J'ai ainsi pris conscience, dès le plus jeune âge, de l'immense sacrifice de nos combattants, qui ont aimé la France au point de lui sacrifier leur vie. Originaire des collines de l'Artois, dans le Pas-de-Calais, j'habitais à quelques mètres de la gigantesque nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette. Je voyais quotidiennement les stigmates laissés par la Première Guerre mondiale. Ces souvenirs sont ceux d'un enfant qui a trouvé l'ancrage de ses valeurs républicaines au contact des anciens, qui se sont battus pour que nous puissions vivre libres. Aussi, je suis particulièrement soucieuse, en pleine crise sanitaire, de protéger nos libertés fondamentales personnelles. Mes chers collègues, les années précédentes, je vous avais fait part de mes profondes inquiétudes sur les crédits de la mission « Anciens combattants, Certes, je constate, cette année, une légère amélioration, mais le sentiment patriotique se dégrade dans une partie de notre jeunesse, la connaissance de l'histoire régresse et la tentation populiste grandit. À vrai dire, ces symptômes, nous les connaissons tous. Personnellement, ils m'inquiètent au plus haut point, car je les ai constatés sur les bancs de l'université, auprès de mes étudiants. C'est une évidence encore plus grande dans les classes de collège et de lycée. L'amour de la France, ça ne se décrète pas- vous en conviendrez, mes chers collègues -, il faut le susciter. Si ces valeurs indispensables à la vitalité de la Nation déclinent, c'est en raison d'une transmission qui ne s'opère plus correctement. Les incivilités constatées dans les classes, lors des cérémonies consacrées au professeur Samuel Paty, ont été dénombrées par le ministère de l'éducation nationale et elles ont été révélées ce matin sur les antennes. Il faut assurer la transmission des valeurs républicaines aux jeunes générations et souligner le sens de la loi égale pour tous. La connaissance du sacrifice consenti par nos anciens combattants doit permettre de comprendre le monde actuel. Je tiens à rendre hommage aux nombreux bénévoles des associations d'anciens combattants, notamment ceux du Souvenir français. Chaque année, de façon totalement désintéressée, ils vont dans les classes des écoles, des collèges et des lycées, partout où l'éducation nationale veut bien les accueillir. Leur témoignage est précieux pour nos enfants, souvent émus par ces rencontres. Ces bénévoles sont des passeurs de mémoire. Absolument ! Les crédits dédiés au programme « Liens entre la Nation et son armée » sont assurément un excellent moyen de faire face à la crise de la citoyenneté. Par ailleurs, j'attire votre attention sur l'amendement de ma collègue Brigitte Micouleau ; nous sommes plusieurs à l'avoir cosigné. Il s'agit d'un amendement de bon sens, visant à réparer une injustice faite aux supplétifs civils de droit commun pendant les conflits d'Afrique du Nord. Ils ne sont plus du Nord. Ils ne sont plus que vingt-cinq à ce jour ; c'est bien peu ... Les supplétifs civils, les harkis, et tous ceux qui ont souffert à un moment de leur vie au nom de la France et pour la France doivent être respectés et reconnus. Il n'y a pas de fatalité en politique. Notre volonté commune est de résoudre cette crise de la citoyenneté qui traverse notre pays. Nous devons nous donner tous les moyens pour réussir. Sur ces travées, nous voulons tous que les jeunes Français aiment leur pays comme nous l'aimons. Pour cela, la France doit avant tout se réconcilier avec son histoire et être fière de tous ses anciens combattants, en leur donnant la reconnaissance qu'ils méritent. La parole est à Mme la ministre

de la République, auquel nous devons des évolutions sociétales majeures, une modernisation du pays et un engagement européen remarquable, au jeune homme de 18 ans qui s'engagea de façon déterminée, à l'été 1944, dans la Première armée française du général de Lattre de Tassigny. Il participa aux combats de la libération du sud-est de la France et poursuivit les combats jusqu'en Autriche. Après huit mois de campagne, il fut décoré de la Croix de guerre 1939-1945. Nous ne pouvons que saluer sa mémoire et cet engagement fort pour la France, dès ses jeunes années. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter ce budget, celui du lien armée-Nation, du lien armée-jeunesse, du monde combattant et de la mémoire. Je sais que vous y êtes attachés et je vous remercie de la qualité des interventions que je viens d'entendre. Avec raison, vous développez ce lien, sur tout le territoire, avec le monde combattant et ses associations.

en diminution de 3 %, en raison de l'attrition naturelle du nombre de ressortissants, est doté de 2 milliards d'euros. Néanmoins, il maintient l'ensemble des dispositifs de reconnaissance, tous les droits et dispositifs fiscaux des anciens combattants et de leurs ayants droit, des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme. Nous y ajoutons des mesures d'amélioration et d'équité, souhaitées par nombre d'associations. Pour nos anciens combattants, notre projet de budget applique d'abord toutes les évolutions que nous avons décidées ensemble depuis 2017. depuis 2017. Je rappelle à ceux qui trouvent que cela ne va pas assez vite, voire ne va pas du tout, que nous avons décidé l'octroi de la carte du combattant aux militaires déployés en Algérie

puisque près de 40 000 cartes ont été délivrées, ce qui est remarquable. Autre exemple : le fonds de solidarité dédié aux enfants d'anciens harkis, doté de 7 millions d'euros, continue de monter en puissance. Nous avons élargi ses conditions d'accès et nous avons pu constater, sur le terrain, l'utilité de ce dispositif et les projets très concrets qu'il finance.

PLF traduit les engagements de ce contrat, avec une subvention de fonctionnement de 56 millions d'euros. Un certain nombre de chantiers de modernisation et de simplification se poursuivront, comme je m'y étais engagée auprès

L'Institution nationale des Invalides- une belle institution -bénéficiera d'une subvention de fonctionnement de 12 millions d'euros et d'une dotation d'investissement de 3,7 millions d'euros, afin de pouvoir démarrer, avant la fin de l'année, la construction des infrastructures qui contribueront à la création du nouveau projet médical, indispensable à nos blessés.

Edgard Tupët-Thomé, Pierre Simonet et, voilà quelques jours, Daniel Cordier -, laissant le flambeau à Hubert Germain. Plus que jamais, nous devons maintenir cette mémoire vive, portée par l'Ordre de la Libération et être attentifs à ce que les crédits affectés à cet organisme soient à la hauteur de nos ambitions mémorielles.

C'est un signe fort, à l'heure où nous avons devant nous les défis liés à la transmission de la mémoire combattante, pilier de nos valeurs républicaines, de l'identité et de la cohésion nationale. Ces crédits permettront de faire face aux besoins d'entretien et de rénovation des nécropoles et de nos dix hauts lieux de mémoire et de financer des cérémonies et des actions éducatives. Nous poursuivrons également notre soutien à la structuration du tourisme de mémoire, enjeu de vitalité sur nos territoires- je sais que vous y êtes sensibles. L'année 2021 sera, en grande partie, consacrée à la mémoire des premiers résistants, notamment ceux de nos outre-mer, et à celle des opérations extérieures, par exemple les trente ans de l'opération Daguet au Koweït. J'ai également souhaité que soit lancée une réflexion sur l'évolution de nos modes de transmission, car, si nous avons dû nous adapter à la crise sanitaire et développer et déployer des outils

La Journée défense et citoyenneté a dû être adaptée aux conditions sanitaires : des séances entièrement numériques ont été mises en oeuvre ces dernières semaines.

afin de pouvoir les dispenser aux jeunes Français à l'étranger. Le service militaire volontaire (SMV) a fait la démonstration de son efficacité avec d'excellents résultats d'insertion. Il a été évalué-

vous annoncer qu'une agrafe « essai nucléaire » pour la médaille de la défense nationale sera créée. Cette décoration honorifique, cette reconnaissance, sera accessible à tous les militaires et personnels civils qui ont participé aux essais nucléaires de notre pays entre 1960 et 1996. 1996. Mesdames, messieurs les sénateurs, ce budget porte sur des sujets éminemment d'actualité : il est celui de la transmission pour l'unité nationale dans les épreuves et de la résilience dans les crises. Je vous remercie de le voter avec enthousiasme.

Compte tenu de l'engagement envers la Nation, de l'âge et de la fragilité des personnes bénéficiaires de la retraite du combattant, il importe de procéder à une revalorisation régulière de l'indice, comme cela avait été fait entre 2007 et 2012. Cela est d'autant plus nécessaire que l'année 2020 a vu l'accroissement de la paupérisation de la population, en particulier des retraités anciens combattants, pour lesquels les sources de revenus sont déjà très limitées. La revalorisation aurait lieu au 1 juillet 2021, pour un coût de 7 millions d'euros, le coût en année pleine s'établissant à 18 millions d'euros.

dégager un million d'euros pour maintenir l'ouverture du droit à percevoir une retraite du combattant à 60 ans pour les titulaires de la carte du combattant domiciliés en outre-mer. À l'instar

La carte du combattant donne droit à la perception d'une retraite du combattant à 65 ans, sauf dans certains cas très particuliers, tenant compte de la situation sociale ou d'invalidité des titulaires de cette carte.

En l'état, le vote de l'amendement n'aurait pas d'effet concret, puisque la base légale permettant d'accéder à la retraite du combattant à partir de 60 ans pour les domiciliés en outre-mer n'existe plus- un amendement

De plus, vous le savez, un monument aux morts pour la France en opérations extérieures a été inauguré le 11 novembre 2019. Vous pouvez le constater : la mémoire des combattants est, d'ores et déjà, honorée par la Nation.

est à Mme Laure Darcos. Je défends cet amendement au nom de ma collègue Brigitte Micouleau. Il s'agit de traiter la situation des membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun. Il serait juste qu'ils puissent bénéficier d'une aide d'un montant de 4 150 euros pour solde de tout compte, afin de réparer, autant que faire se peut, le comportement injuste de l'administration à leur égard

aux présidents de commission, afin qu'ils soient informés de cette évolution. Je vous invite, si vous avez des doutes, à consulter la directrice générale de l'ONAC-VG. Je peux vous assurer que nous sommes très attentifs à ces dossiers.

Au regard du temps restant et dans la mesure où il serait difficile d'entamer ce bloc de missions avant minuit, nous pourrions d'ores et déjà décider, en accord avec la commission des finances, les commissions concernées et le Gouvernement, d'en reporter l'examen à demain, samedi 5 décembre matin.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,

En effet, pour le sport, la jeunesse et la vie associative, le coup est rude et ses effets se poursuivent. Les pratiques sportives demeurent interrompues sur l'ensemble du territoire. La jeunesse subit de plein fouet des restrictions nécessaires, mais douloureuses, tandis que la vie associative doit se réinventer à l'heure de la « distanciation sociale Pour autant, ces trois axes sont plus que jamais indispensables pour réaffirmer une cohésion nationale ébranlée. Je retiendrai deux points généraux de présentation. Pour 2021, les crédits proposés pour la mission connaissent une hausse de 12,5 % par rapport à l'année précédente. Il s'agit non pas d'une réponse à la situation actuelle, mais bien d'une tendance de fond, qui s'explique essentiellement par le service national universel (SNU) et la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. ces deux postes de dépenses était prévue, mais à défaut de trajectoire budgétaire actualisée, rien n'indique comment la soutenabilité de la mission, dont les crédits ont été multipliés par 2,7 depuis 2015, sera assurée. Cette progression s'accompagne d'une concentration exceptionnelle des dépenses portées par la mission, qui en affecte la capacité de pilotage. Trois dispositifs représentent les trois quarts de ses crédits : la subvention à l'Agence nationale du sport (ANS), les politiques de l'engagement de la jeunesse- service civique et service national universel -et les Olympiades de 2024. L'analyse des crédits est toutefois altérée cette année, en raison de la multiplication des vecteurs budgétaires : les collectifs budgétaires, le projet de loi de finances, mais aussi la mission dédiée au plan de relance. La mise en oeuvre de celui-ci, dont les crédits sont concentrés sur une mission spécifiquement créée, viendra compléter le soutien aux politiques de la mission, à hauteur de 437 millions d'euros en crédits de paiement. Cependant, plus de 80 % de ce montant résulte de la comptabilisation des dépenses tendant à augmenter de 100 000 le nombre de jeunes en service civique en 2021, dont la labellisation « relance » me surprend quelque peu. Madame la secrétaire ne faut-il pas s'interroger sur les capacités d'absorber un tel contingent supplémentaire sans que la qualité des missions proposées soit rognée ? Par ailleurs, la quatrième loi de finances rectificative pour 2020 a prévu d'importants crédits pour la mission, qu'il nous faut prendre en compte. Le soutien à la vie associative a été abondé de 35 millions d'euros. Pour le sport, plus de 100 millions d'euros ont été alloués aux clubs pour compenser les pertes de billetterie et, sur l'initiative du Sénat, la réserve des crédits a finalement été dégelée.

67 millions d'euros de décaissements, et du relèvement du plafond de la fiscalité affectée à l'Agence nationale du sport. Je m'en réjouis, car cet effort est indispensable pour soutenir le secteur du sport. Pour autant, je reste prudent, car le relèvement du plafond de la fiscalité affectée à l'ANS prend acte du dynamisme marqué du produit de la taxe Buffet. Or celui-ci s'explique essentiellement par le nouveau contrat de diffusion du championnat de football professionnel, dont chacun ici aura suivi la chronique juridique qui s'est engagée depuis la rentrée. En cas de nouvel appel d'offres, lequel est loin d'être exclu, rien ne garantit que le montant du contrat soit équivalent, ce qui pourrait porter les recettes fiscales sous le plafond prévu en 2021. En privilégiant le relèvement du plafond à une majoration de la subvention versée à l'Agence nationale du sport, le Gouvernement transfère donc le risque vers le mouvement sportif. Madame la ministre, pouvez-vous nous rassurer et nous garantir que, si le rendement de la taxe Buffet est moindre qu'escompté, des crédits budgétaires seront débloqués pour compenser ? Le deuxième point concerne le service national universel. En 2020, 30 millions d'euros étaient prévus, pour un objectif de 20 000 jeunes, soit un coût moyen par jeune de 1 500 euros. La crise sanitaire aura toutefois marqué un coup d'arrêt. L'année 2021 doit permettre de reprendre la mise en oeuvre de ce dispositif, pour un objectif de 25 000 jeunes. Mais, entretemps, les prévisions ont été quelque peu revues

L'an dernier, nous avions adopté un mécanisme de fléchage d'une partie des avoirs des comptes inactifs revenant à l'État vers le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA).En 2021, ce sont 17,5 millions d'euros qui pourraient ainsi lui être versés. Dans ces conditions, la commission

Monsieur le président, madame la ministre, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, en juin dernier, notre commission avait affirmé que « la crise que connaît le secteur du sport était profonde et durable » et regretté qu'à cette date « aucun plan de relance digne de ce nom n'ait été présenté et mis en oeuvre ». Il aura fallu attendre huit mois pour que le Gouvernement prenne la pleine mesure du choc, auquel le mouvement sportif est confronté depuis mars dernier, et réagisse, au travers d'annonces successives, à mesure que la situation du secteur se détériorait. Une première étape, trop modeste, avait consisté en la mise en place, en juin 2020, d'un fonds de solidarité de 15 millions d'euros, afin de soutenir les petites associations sportives. Ce fonds est reconduit en 2021. La présentation du PLF 2021 a constitué une deuxième étape plus significative, avec, d'une part, une hausse des moyens de l'Agence nationale du sport et, d'autre part, la mise en place d'un plan de soutien au secteur du sport. L'ANS bénéficiera de la totalité du produit de la taxe Buffet, soit 74,1 millions d'euros, ce qui représente une hausse globale de 34,1 millions. Nous nous réjouissons du déplafonnement de cette taxe, lequel constituait une revendication ancienne de la commission de la culture. L'annonce d'une enveloppe de 122 millions d'euros sur deux années, portée à 132 millions à l'issue de l'examen du budget à l'Assemblée nationale, a constitué une autre annonce importante. Nous avons été nombreux à partager le sentiment exprimé par le mouvement sportif en octobre dernier que le plan de relance n'était pas équilibré, puisque seulement 21 millions d'euros étaient destinés aux clubs. Afin de répondre aux conséquences du huis clos dans les enceintes sportives, le Gouvernement a annoncé la création d'un fonds de compensation des pertes de billetterie, doté de 110 millions d'euros. Outre que cette somme ne représentera qu'une petite partie des pertes des quelque 150 structures qui peuvent y prétendre, nous aurions souhaité que le fonds perdure au moins jusqu'à juin 2021, puisqu'il est peu probable qu'un fonctionnement normal soit rétabli d'ici là. La troisième étape a été marquée par plusieurs annonces faites par le Président de la République le 17 novembre dernier, dont la création du Pass'Sport. Ce dispositif, doté de 100 millions d'euros, devrait voir le jour en 2021 afin d'aider les publics les plus fragilisés à accéder à la pratique sportive. Je propose depuis deux ans la création d'un dispositif similaire. Je rappelle qu'il doit être articulé avec les initiatives des collectivités territoriales afin d'atteindre un montant d'environ 300 euros, permettant de financer le coût de la licence, la cotisation aux clubs ou divers

En conclusion, ce budget présente de vraies avancées, notamment sur la préparation des jeux Olympiques, le laboratoire de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et le maintien des conseillers techniques sportifs (CTS) dans le giron de l'État. Toutefois, les mesures de soutien au secteur du sport auront été trop tardives, ce qui n'a pas permis d'en assurer le financement complet dans le PLF pour Notre commission a émis un avis favorable sur l'adoption des crédits, non sans insister sur la nécessité de clarifier au plus vite le financement des annonces du Président de la République et de prolonger les dispositifs au moins jusqu'au printemps 2021. La parole est à M. applaudissements,

Toutefois, le doublement du budget consacré au service national universel (SNU) explique en grande partie cette augmentation. Or la commission a exprimé de nombreuses réserves sur ce dispositif. Le coût en est élevé : 2 300 euros par jeune, contre 1 000 à 1 500 euros évoqués lors de sa création.

Ainsi, ce sont 60 millions d'euros, soit 10 % des crédits du programme, qui sont consacrés à un dispositif aux contours flous, déployé sans concertation et dont la réalisation en 2021 est incertaine. Dans le même temps, les moyens alloués aux associations fortement touchées par la crise sont trop modestes. Pour rappel, 66 % des associations ont complètement suspendu leurs activités, 55 000 déclarent ne pas pouvoir maintenir les salaires et les déclarations d'embauche sont en chute de 45 %. Lors de la campagne du FDVA de 2020, le nombre de demandes de subvention était deux fois plus nombreux que celui des dossiers retenus, et les montants alloués deux à trois fois inférieurs aux demandes. Entretemps, la crise sanitaire et économique est arrivée et, avec elle, les difficultés financières pour les associations. Je souhaite également évoquer la situation des acteurs du tourisme social. Ces derniers ont également été très fortement touchés par la crise. La totalité des classes vertes a été annulée entre mars et juin 2020. Les colonies de vacances, malgré le dispositif Vacances apprenantes, ont connu un taux de remplissage faible pendant les vacances d'été. Dans le cadre du PLFR 4, 15 millions d'euros venant des crédits non utilisés du SNU ont permis de soutenir les acteurs des colonies de vacances et des séjours pour enfants. Est-ce suffisant ? Je crains que non. Actuellement, le taux de réservation est de 80 % inférieur à celui de l'année dernière à la même date. Le Gouvernement souhaite promouvoir la cohésion nationale et la citoyenneté, notamment à travers le SNU. la citoyenneté se construit avant 16 ans, l'école, le temps périscolaire et les colonies de vacances, qu'il est urgent d'accompagner et de renforcer. Je conclurai mon propos, en évoquant la mission « Plan de relance ». La commission a salué les 609 millions d'euros en faveur de la jeunesse et des associations qui sont inscrits dans cette mission- je tenais à le préciser. Certaines mesures sont ambitieuses. Je pense aux 100 000 nouvelles missions de service civique qui devront être créées. Cela nécessite la mobilisation de tous, mais aussi une vigilance accrue dans le contrôle de la qualité des missions. Je souhaite également que les jeunes des territoires ruraux ne soient pas oubliés dans ce dispositif. je regrette l'inscription d'un certain nombre de mesures dans cette mission qui augurent d'un caractère conjoncturel du surcroît d'attention du Gouvernement en faveur de la jeunesse et la vie associative.

ministre, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, il a fallu beaucoup de temps pour que le Gouvernement prenne en compte le choc provoqué par la crise sanitaire sur le mouvement sportif.

Les mesures dont on pourrait se réjouir ne sont pas toutes budgétées dans ce PLF, y compris celles que vous venez de détailler voilà quelques heures, madame la ministre. Ainsi, si je salue bien évidemment le déplafonnement de la taxe Buffet affectée à l'Agence

Au-delà de la crise sanitaire, nos inquiétudes s'accroissent sur le modèle sportif qui se dessine, mesure après mesure. C'est désormais un groupement d'intérêt public (GIP) qui définit la politique sportive de la France. La mobilisation a empêché le transfert des CTS vers les fédérations, mais leurs effectifs continuent de fondre. L'Agence française de lutte contre le dopage doit faire toujours plus sans moyens supplémentaires et notre parc d'équipements vieillit inexorablement. Les crédits affectés à la préparation des jeux Olympiques de Paris ne sauraient masquer cette situation. Pourtant, la pratique sportive est préconisée. Elle est même indispensable pour lutter contre les comorbidités, facteur aggravant du covid. Les clubs ont et auront aussi un rôle décisif à jouer pour retricoter le lien social, tellement distendu ces temps-ci, à condition de pouvoir rebondir. Ce budget ne le permettra pas. Les crédits affectés à la jeunesse et à la vie associative paraissent eux aussi bien dérisoires dans le contexte actuel. Nous avons conscience que la mission examinée aujourd'hui ne résume pas à elle seule l'ensemble

Quoi que l'on pense du SNU, il ne saurait être la priorité du moment. Le séjour de cohésion, qui constitue la première phase du dispositif, n'a pas eu lieu au printemps dernier. Et pour cause ! Au reste, nul ne sait, si les missions d'intérêt général qui en composent la deuxième phase verront le jour,

Celui-ci bénéficiera d'environ 15 millions d'euros issus des comptes bancaires inactifs- enfin ! Toutefois, chacun sait déjà que ce sera insuffisant. La création de nouveaux contrats de service civique peut répondre en partie à la situation d'urgence, mais il faudra veiller aux abus en termes d'emplois déguisés, inhérents au dispositif même et dont les risques peuvent se trouver renforcés par la situation de fragilité que connaissent les différents acteurs qui recrutent ces services civiques.

Quant aux parcours emploi compétences, les deux cents maires mobilisés pour alerter sur le risque de décrochage des quartiers populaires les jugent notoirement insuffisants. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ces budgets.

de rendre opérationnelles, sur tout le territoire, des ambitions empreintes d'une véritable grandeur, la crise sanitaire et sociale sans précédent que nous traversons aurait dû être l'amorce d'une véritable approche pragmatique et pérenne pour la mission « Sport, jeunesse et vie associative ». Or que constatons-nous ? À la fois beaucoup de temps perdu et la mise en exergue de certaines actions au détriment d'autres, comme en témoignent la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques et le SNU, qui accaparent pratiquement tout, le reste étant renvoyé au plan de relance.

Certes, la perspective de cet événement extraordinaire doit être portée par un programme budgétaire digne de ce nom, et nous saluons bien évidemment cette ligne du Gouvernement. Cependant, n'oublions pas les territoires, qui pâtissent une fois encore du manque d'épaisseur de l'exercice budgétaire, alors même que les champions de demain s'entraînent aujourd'hui dans les territoires, d'où ils doivent émerger.

la situation des bénévoles, dont le renouvellement va poser problème. Le sport français a besoin de ressources supplémentaires pour assurer sa présence sur la durée dans tous les territoires. Les clubs en ont besoin pour anticiper, développer et répondre aux attentes des Français et pour renforcer l'emploi et la formation des éducateurs et des entraîneurs. Ils en ont besoin pour investir, aux côtés des collectivités locales, dans des équipements sportifs qu'elles détiennent à près de 85 %, mais qui, aujourd'hui, vieillissent et sont insuffisants et inadaptés. Le sport professionnel est lui aussi en souffrance. C'est toute une économie qui est en danger, avec l'arrêt des compétitions ou les rencontres à huis clos, qui font chuter les recettes de billetterie et révèlent de grandes disparités entre les disciplines. Or le monde sportif a un rôle crucial à jouer en faveur de l'éducation, de la cohésion sociale et de l'insertion, mais aussi de la santé et du développement durable. À ce titre, nous devons pleinement soutenir ce secteur, fortement touché par la crise. Les 34 millions d'euros de taxes affectées supplémentaires suffiront-ils ? Les 120 millions d'euros sur deux ans du plan de relance, dont une grosse part sera dédiée à la rénovation énergétique des équipements sportifs, suffiront-ils à aller chercher les trois millions de pratiquants ? le plan de relance, qui apparaît plus comme un plan de rattrapage, montre bien les insuffisances du projet originel, puisqu'il contient de nécessaires rallonges financières, en particulier à destination du monde associatif sportif local. Au final, le budget du ministère chargé des sports semble en hausse en 2021, la période actuelle, que nous pouvons qualifier d'extraordinaire, aurait dû pousser le Gouvernement à s'engager

qui, soit dit en passant, n'a jamais retrouvé son niveau du temps de la réserve parlementaire- environ 50 millions d'euros -permettra-t-il de relever les défis ? Les associations, dont le dévouement sans faille doit être souligné, sont en péril. Certes, les associations employeuses ont pu bénéficier des mesures développées pour les entreprises, mais toutes les autres petites associations, dont la plupart ne peuvent compter que sur le bénévolat, doivent plus que jamais être accompagnées. Leurs pertes financières sont importantes, voire abyssales, du fait notamment de l'annulation de la quasi-totalité des événements, mais aussi en raison d'une reprise plus que chaotique des activités. C'est la raison pour laquelle, comme nombre

Compte tenu du contexte et de la faible portée du dispositif à l'heure actuelle, n'est-il pas disproportionné de doubler les crédits du SNU, pour les porter à plus de 60 millions d'euros, quand ils ne répondent pas aux attentes de la jeunesse ? L'enjeu d'aujourd'hui est de répondre à la précarité. Voilà l'urgence Pour conclure, même si elles sont différées, je veux saluer l'ensemble des mesures pour le sport annoncées tout récemment par le Gouvernement : enveloppe de quelque 100 millions d'euros pour le Pass'Sport, compensation des pertes de recettes et de billetterie, mesures d'urgence l'ANS pour soutenir les clubs, etc. Ainsi, si nous avions la possibilité de dissocier, au sein de cette mission, le programme « Sport » du programme « Jeunesse et vie associative », notre groupe voterait pour le premier et s'abstiendrait sur le second. Puisque ce n'est pas le cas et compte tenu du manque de pragmatisme et du

nous sommes [ ...] désemparés par le peu de considération dont nous faisons l'objet alors que nous avons un rôle important à jouer au sein de la Nation. Le plus difficile est d'accepter que le Gouvernement ne s'adresse à nous qu'en cas de problème Tout est dit dans cette phrase, prononcée devant notre commission, voilà quelques jours, par le président du CNOSF. Nous sommes nombreux, madame la ministre, à partager ce constat. Le monde sportif, amateur et professionnel, traverse une crise sans précédent avec un arrêt total ou partiel des activités, une chute du nombre de licenciés, un risque de voir les partenaires publics et privés revoir leur soutien à la baisse, un recul du nombre de bénévoles ; bref, une situation qui inquiète l'ensemble de l'écosystème du sport. Face à cette crise, les crédits inscrits dans le budget pour 2021 sont-ils à la hauteur des besoins ? Pour notre part, nous pensons que non. L'impact de cette crise sanitaire sur le monde sportif est largement sous-estimé par le Gouvernement. Si nous étions dans une année « normale », nous aurions pu dire que le budget que vous nous proposez pour 2021 va dans le bon sens avec une augmentation de 8 millions d'euros, à laquelle il faut ajouter les 34 millions d'euros liés au déplafonnement de la taxe Buffet que nous appelions de nos voeux. appelions de nos voeux. Mais, voilà, nous ne sommes pas dans une période normale. Si nous pouvons souligner la hausse du programme 350 consacré aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, cette évolution est normale et attendue. Elle concerne la construction des villages des athlètes et des médias, qui seront transformés en logements. Par ailleurs, je tiens à souligner que l'État n'a toujours pas honoré sa contribution de 80 millions d'euros au comité d'organisation Paris 2024 au titre des jeux Paralympiques

De plus, il existe un réel besoin de porter des actions de sensibilisation et d'information sur le terrain auprès des éducateurs et des licenciés sur des enjeux majeurs comme la lutte contre le racisme, les violences sexuelles, le dopage, l'homophobie, les dérives religieuses et autres problèmes qui gangrènent le sport dans notre pays. notre inquiétude porte sur les difficultés financières de l'Insep, qui a considérablement entamé sa trésorerie et fait une croix sur des opérations d'entretien et d'investissement pour compenser sa perte de recettes. Enfin, comme l'a rappelé notre rapporteur, nous constatons la situation financière tendue de l'Agence française de lutte contre le dopage face à l'accroissement de ses missions. Je tiens cependant à saluer la mesure nouvelle de 3,5 millions d'euros visant au financement des maisons sport-santé, si des interrogations demeurent sur la formation des encadrants et, surtout, sur le remboursement des séances de pratiques. Sur les autres missions, vos propositions ne sont pas satisfaisantes.

Le Président de la République a annoncé 400 millions d'euros, mais nous savons que ces chiffres ne reflètent pas la réalité : une partie de cette somme consiste à recycler les dispositifs adoptés dans le PLFR 4 et le PLFSS à hauteur de 212 millions d'euros, le reste n'étant toujours pas budgété. Ce n'est pas très sérieux. C'est la raison pour laquelle nous présenterons des amendements visant à apporter un réel soutien au sport, aussi bien amateur que professionnel. Je me permets de rappeler le vote de 4,7 millions d'euros sur le budget sport pour 2020, que le Gouvernement souhaitait

un soutien à l'apprentissage de la natation durant le parcours scolaire de 5 millions d'euros. Nous avons créé un fonds de soutien doté de 10 millions d'euros pour les associations sportives agissant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, où, là encore, les acteurs se sentent abandonnés et oubliés par l'État. également adopté un nouveau dispositif sur le droit à l'image. Nous avons donc pleinement joué notre rôle pour soutenir le sport. Désormais, madame la ministre, nous avons besoin de savoir si, oui ou non, vous soutiendrez ces nouveaux financements devant les députés.

Le sport amateur et professionnel, les petits comme les grands clubs, tous font face à cette crise. Permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour les bénévoles, qui font vivre en grande partie la pratique du sport et nos associations dans notre pays. Sans eux, sans leur dévotion rien ne serait possible. La chute du nombre d'adhérents, et certainement des bénévoles, aura des conséquences. Nous devrons les soutenir. La crise frappe de plein fouet le secteur associatif. De nombreuses transformations sont à l'oeuvre dans les structures traditionnelles. Les moyens Les moyens alloués aux différents programmes sont donc cruciaux, au même titre que le plan de relance et les annonces du Président de la République du 17 novembre dernier, sur lesquelles je terminerai mon propos.

Depuis trois ans, nous constatons que le budget du programme « Sport » se renforce grâce à l'objectif des JO 2024. Rendez-vous incontournable du sport de haut niveau mondial, ces jeux constitueront un atout et une vitrine pour notre pays. Ils doivent aussi l'être pour le sport et sa pratique sur notre territoire. raison pour laquelle, comme notre groupe l'an dernier, je plaide pour des financements importants dans les domaines hors jeux Olympiques. La hausse de plus de 20 % des crédits dans le programme « Sport » est encourageante, mais les enjeux restent fort nombreux. concerne l'Agence nationale du sport. Nous avions l'an dernier souligné l'importance de sa création et de ses missions pour nos territoires et nos concitoyens. Son financement, notamment grâce au plan de relance, enregistre une hausse importante ; cela va dans le bon sens. La vie associative dans notre pays est un élément essentiel de cohésion nationale, de lien social et de vie en commun. L'an dernier, nous avions signalé que le Fonds pour le développement de la vie associative était trop peu doté. Cette année encore, malgré des améliorations, la dotation semble toujours insuffisante. insuffisante. Le sport était le grand oublié du plan de relance. Son enveloppe de 122 millions d'euros est bien loin des 2 milliards d'euros consacrés à la culture. Loin d'opposer les deux, je veux simplement rappeler l'importance du sport pour la vie des Français, ses missions d'éducation et de santé publique. En réponse aux appels à l'aide lancés par le milieu du sport, le Président de la République a annoncé 400 millions d'euros d'aides supplémentaires. d'aides supplémentaires. C'est une bonne nouvelle, malgré un manque de lisibilité et des moyens éclatés dans plusieurs mécanismes : plan de relance, exonérations de cotisations sociales patronales prévues dans le PLFSS, fonds de solidarité pour les clubs les plus touchés par la crise ou encore fonds de compensation pour la billetterie ... Déjà des craintes s'expriment sur de possibles dépôts de bilan. Les aides sont pour beaucoup en deçà des espoirs créés lors de ces annonces. La réaction doit être rapide. Nous devons trouver des aménagements, notamment pour les jauges. Dès janvier prochain, elles doivent être calibrées en fonction des infrastructures. Nous regrettons que cela n'ait pas déjà été fait. L'année qui arrive nécessitera de nouveaux ajustements, et nous devrons être au rendez-vous. La jeunesse, la vie associative, le sport font la cohésion de notre pays et la France de demain. Nous avons le devoir de réussir.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, comme tous les crédits que nous avons eu à examiner dans la deuxième partie de ce projet de loi de finances, ceux de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » s'inscrivent dans le contexte de la pandémie globale, qui met à l'épreuve notre système dans son ensemble. L'activité sportive, qu'elle soit pratiquée en amateur ou en professionnel, subit toujours les effets des différents confinements, et les perspectives restent très sombres. Entre les stades vides et le conflit entre la ligue et Mediapro, le football professionnel est dans une situation extrêmement alarmante. Cependant, la situation de l'ensemble des fédérations sportives est tout aussi préoccupante. De nouvelles annonces ont été faites par le Gouvernement, mais des amendements que nous examinerons dans quelques instants proposeront des pistes un peu plus ambitieuses pour leur venir en aide. Les associations, notamment celles oeuvrant pour la solidarité, se sont révélées être des acteurs de première ligne pour amortir les effets de la crise. engagées dans la lutte contre la précarité ont effectué un indispensable travail de soutien envers les plus fragiles, alors que nous étions tous confinés au printemps. Ce travail a continué jusqu'à maintenant, tant les besoins sociaux ont explosé. Il faut le reconnaître, le Gouvernement s'est mobilisé pour les soutenir à travers le plan de relance. Ce sont ainsi plus de 609 millions d'euros qui ont été mobilisés pour soutenir le service civique, avec 100 000 missions supplémentaires, pour accompagner la création d'emplois dans le sport, pour favoriser la transition numérique des acteurs, sans compter les diverses mesures de soutien aux associations le Fonds pour le développement de la vie associative ou la rénovation des équipements. Cependant, ce soutien est par nature exceptionnel et limité dans le temps. Quand on regarde les crédits budgétés, on constate une stabilité des montants alloués à la plupart des dispositifs. En effet, la hausse de 12,5 % des crédits de paiement de la mission s'explique principalement par l'augmentation des fonds pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et pour le service national universel. pour faire des jeux Olympiques et Paralympiques un événement planétaire exemplaire en matière environnementale. Il conviendra d'y être extrêmement vigilant. Les enjeux climatiques nécessitent la mobilisation de toutes et tous, y compris et surtout les grands événements. Aujourd'hui, le budget augmente très fortement, mais reste toutefois dans les clous des engagements pris. Nous devons rester très attentifs à cette question, tant les coûts ont explosé à des niveaux pharaoniques par le passé pour tous les pays organisateurs, sans exception.

un simple prélude au milliard et demi d'ores et déjà annoncé -, et ce alors même que l'expérimentation initiée l'année dernière a été mise à l'arrêt en raison de la pandémie, nous apparaît totalement injustifié au regard de la conjoncture. Sur le fond, nous nous opposons à l'existence même du service national universel. Il existe déjà un service civique qui qui vient de fêter ses dix ans et qui reçoit l'adhésion quasi unanime de tous ses acteurs et de ses volontaires. Il incarne bien mieux l'esprit de mobilisation de la jeunesse que ce service national dont les uniformes et oripeaux d'autorité républicaine cachent bien mal l'absence de sens profond. Il est donc d'autant plus désolant de constater que le service civique- hormis dans le plan de relance -ne voit pas ses crédits augmenter sur le long terme. Nous nous félicitons naturellement des mesures exceptionnelles en direction du sport et de la jeunesse, mais nous regrettons la construction de ce budget, qui privilégie un soutien ponctuel plutôt qu'une dynamique de long terme sur les dispositifs

jeunesse et vie associative » dans le budget pour 2021 est inédit. En effet, il représente près de 1,4 milliard d'euros en crédits de paiement, soit une progression de 12,5 par rapport au PLF pour 2020. Oui, ce montant est inédit, puisque les crédits alloués à la mission ont presque été multipliés par trois depuis 2015 ! En somme, le budget pour 2021 accélère cette montée en charge pour l'ériger au rang de priorité, et il convient de le saluer. Il faut par ailleurs ajouter à ces crédits ceux du plan de relance, qui comprend pas moins de 437 millions d'euros en crédits de paiement, dont 67 millions d'euros pour le sport et 370 millions d'euros pour la jeunesse et la vie associative. Au bout du compte, mes chers collègues, le budget pour 2021 pour le sport, la jeunesse et la vie associative est sans précédent. Pour le sport, le budget pour 2021 confirme une montée en puissance importante du programme 350 dédié au financement des JO de Paris 2024 234 millions d'euros lui sont alloués, soit deux fois plus qu'en 2020. Le plan de relance, quant à lui, ouvre une enveloppe de 122 millions d'euros sur deux ans qui viendra abonder les moyens de l'Agence nationale du sport, dont les crédits augmentent en 2021 de près de 30 % pour s'établir à 365 millions d'euros. Ces moyens supplémentaires vont d'abord soutenir les clubs et les fédérations, qui ont été très affectés par l'arrêt de leurs activités au printemps dernier et dont la reprise est difficile depuis le mois de septembre. des crédits de l'Agence nationale du sport issus du plan de relance sera d'ailleurs consacrée à la création d'un fonds de compensation pour amortir les pertes des fédérations sportives en termes de licences. Je salue, madame la ministre, les mesures avez annoncées avec le Président de la République, notamment la création du Pass'Sport. Par ailleurs, permettez-moi de rappeler qu'en deuxième lecture du PLFSS à l'Assemblée nationale un amendement du Gouvernement a permis aux clubs sportifs professionnels de moins de 250 salariés de bénéficier du dispositif d'exonération de cotisations sociales patronales hors retraite complémentaire et d'aide au paiement des cotisations dues en octobre, novembre et décembre. Ce dispositif représente un effort de 105 millions d'euros destiné aux clubs sportifs professionnels, qui n'ont quasiment plus de recettes du fait des restrictions de jauge,

les associations, dont les activités ont été très touchées par la crise sanitaire et qui constituent un pilier de la solidarité dans notre pays. Ainsi, le Fonds pour le développement de la vie associative bénéficiera, à partir de 2021, d'un abondement annuel venant des comptes inactifs des associations tombées en déshérence- il faut saluer cette hausse de moyens.

Dans ce contexte, on ne peut que se réjouir de l'augmentation de 12,5 % de ses crédits de paiement et de 5,5 % de ses autorisations d'engagement pour 2021. Ainsi, 2021. Ainsi, les moyens alloués au sport sont renforcés, notamment pour répondre à l'accélération des chantiers en vue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. En outre, si l'on y agrège le plan de relance, hors olympiades, c'est une hausse de 21 %, soit un effort sans précédent qui était plus que nécessaire compte tenu de l'ampleur de l'impact de la pandémie. En effet, si les compétitions et matchs ont pu reprendre, la situation est très critique pour le sport professionnel. La jauge a oscillé entre restriction partielle et interdiction totale : un coup de massue pour les clubs les plus dépendants des « recettes stade stade ». La quasi-disparition des recettes de billetterie et le maintien de règles sanitaires extrêmement strictes ont rendu l'équation compliquée pour les organisateurs d'événements sportifs et les clubs.

Le football est un sport très populaire, très fédérateur au moment des grands événements. Il serait difficile de laisser le secteur s'effondrer. Mais de quelle marge disposent les pouvoirs publics pour encourager, dans les conditions actuelles, la réforme d'un modèle économique économique déjà fragilisé bien avant la crise sanitaire ? L'affaire Mediapro en est, hélas, une illustration, et souligne la prépondérance des droits TV dans les revenus des clubs. Au-delà des événements sportifs, la pratique sportive amateur se retrouve également très affectée. On observe un véritable décrochage sportif. Vous connaissez les chiffres, madame la ministre : selon le Comité national olympique et sportif français, un licencié sur quatre ne s'est pas réinscrit en club pour l'année 2020. alarmant : des structures moins médiatisées se retrouvent dans la difficulté. Je pense à l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique ou encore à la Fédération du sport adapté, qui intéresse les personnes en situation de handicap mental. Ces cas risquent d'affaiblir l'une des politiques prioritaires du Gouvernement, à savoir la promotion de l'accès au sport pour tous. Un véritable plan d'urgence est réclamé par les professionnels, qui souhaitent pouvoir passer le cap de la crise. Il faut absolument soutenir tous ceux qui oeuvrent pour un sport plus inclusif et contribuent ainsi aux fondements de notre pacte républicain. En ce qui concerne la jeune Agence nationale du sport, pourriez-vous nous apporter des garanties, madame la ministre, quant à sa volonté de rétablir les égalités territoriales en matière d'équipements sportifs publics. L'atténuation des inégalités sociales dans le sport passe aussi par le développement des équipements publics. Il faut Il faut donc davantage les encourager, en particulier en milieu rural. S'agissant de l'autre grand volet de la mission, la jeunesse et la vie associative, on observe que la hausse de 6 % des crédits financera en grande partie la montée en charge du service national universel. Beaucoup de nos jeunes concitoyens vont souffrir de la crise économique. Cette situation oblige à la protection des entités qui donnent corps à la cohésion sociale et leur offrent une solution d'attente. Dans cet esprit, je note que le budget tient compte des conséquences de la crise sanitaire en prévoyant de majorer les crédits du Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire, ainsi que ceux des deux fonds de développement de la vie associative. Mon groupe y est sensible, de même qu'au renforcement du service national universel, doté de 32,5 millions d'euros supplémentaires. Le RDSE est en effet attentif à tout ce qui touche à l'engagement citoyen. Je rappelle que notre ancien collègue et président du groupe, Yvon Collin, avait porté la création du service civique, qui attire de plus en plus de jeunes. Mes chers collègues, à l'heure où l'on parle d'une génération « covid » avec un sous-entendu sacrificiel, tout doit être mis en oeuvre pour faire plutôt de cette jeunesse

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,

Mais il s'agit, comme trop souvent avec votre gouvernement, d'un volontarisme de façade ! À travers l'examen de ces crédits, on ne peut que regretter l'absence de réelle inflexion de la politique gouvernementale.

et un renforcement des financements de projets qui ne correspondent pas aux aspirations de la jeunesse, l'exemple le plus frappant étant celui du service national universel, comme cela a déjà été souligné à plusieurs reprises. Le programme 163, c'est 699 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Sur les 39 millions d'euros supplémentaires inscrits, le SNU en accapare 32 millions, la dotation totale du SNU atteignant ainsi 62 millions d'euros. n'a pourtant pas fait la preuve de son utilité avec une redondance des formations et des modalités d'engagement par rapport à d'autres dispositifs. Le service civique, lui, connaît un véritable engouement de la part des jeunes. Ainsi, en cinq ans, le nombre de volontaires a quadruplé 35 000 en 2014 à 145 000 en 2019. Or on observe une stagnation de ses crédits budgétaires. Certes, ce dispositif bénéficie du financement du plan de relance, mais on entend bien qu'il ne s'agit pas de financements pérennes. Je veux maintenant évoquer les associations, dont nul ne peut contester le rôle essentiel de cohésion en ces périodes très difficiles. Les associations subissent de plein fouet les effets de l'épidémie avec des suspensions d'activités pour certaines et un afflux de demandes, bien souvent liées à la désespérance sociale, Pour venir en aide aux associations, qui traversent une crise considérable, aux implications non encore mesurées, il aurait fallu augmenter fortement les moyens du Fonds pour le développement de la vie associative. Mais tel n'est pas le cas. Pour augmenter les crédits du FDVA, on ne peut se contenter des 15 millions d'euros issus des comptes inactifs, mécanisme voté dans la loi de finances pour 2020, même si cette initiative, portée notamment par notre collègue Jacques-Bernard Magner, a permis de dégager des fonds supplémentaires bienvenus.

Le Fonjep permet le développement de l'emploi au sein des associations, démarche extrêmement utile en ces périodes. Nous notons un changement d'orientation politique par rapport au début du quinquennat, qui avait vu la réduction drastique des contrats aidés, erreur politique grave dénoncée sans relâche par notre groupe.

La hausse des crédits du sport se concentre en très grande majorité sur le programme 350 dédié aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024, en particulier pour la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo). Avant même la crise exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés, le sport n'était malheureusement pas accessible à tous, y compris dans le cadre scolaire. Nous sommes très attentifs aux inégalités d'accès à la pratique du sport, en particulier dans les territoires ruraux. La crise sanitaire liée à la covid-19 agit bien évidemment comme un tsunami sur le sport amateur comme sur le sport professionnel. La déstabilisation est générale : le nombre de licenciés sportifs va baisser, parfois même de 20 % à 30 %. La demande de soutien au sport amateur et professionnel est massive face aux conséquences déstabilisatrices de la crise sanitaire. Ainsi, plus de 4 000 clubs de foot ont cessé leur activité, en particulier en milieu rural. Le besoin de financement est donc urgent. Il est urgent aussi de dédier davantage de moyens à la pratique sportive féminine, notamment au foot. Les acteurs du sport professionnel et amateur ont l'impression d'être exclus des priorités de la Nation, comme l'a constaté le président du Comité national olympique et sportif français lors d'une récente audition devant notre commission. Il a chiffré les pertes à près de 1 milliard d'euros. Le Président de la République a récemment annoncé une enveloppe de 400 millions d'euros pour le sport amateur et professionnel, qui s'avère, hélas, trop faible et sous-dimensionnée. Il est urgent de mettre en place la mesure très attendue du Pass'Sport, projet porté depuis de nombreuses années par notre rapporteur pour avis Jean-Jacques Lozach. Ce dispositif permettra d'aider les familles à payer les inscriptions en clubs et l'achat d'équipements sportifs. Une enveloppe de 100 millions d'euros par an est annoncée, mais le flou demeure puisque le Gouvernement ne précise ni la cible ni le nombre de jeunes concernés. Les sénateurs Socialistes, Écologistes et Républicains présenteront tout à l'heure un amendement visant à concrétiser la création de ce Pass'Sport. J'espère que la Haute Assemblée validera ce dispositif. Le budget de la mission « Sport, jeunesse et vie associative au-delà du volontarisme gouvernemental affiché, est en trompe-l'oeil. Il n'est malheureusement pas à la hauteur des énormes difficultés que traverse notre pays. C'est la raison pour laquelle les sénatrices et sénateurs Socialistes, Écologistes et Républicains voteront contre ces crédits. La parole est à la toute jeune

la secrétaire d'État, mes chers collègues, la jeunesse et la vie associative, qui font l'objet du programme 163, sont deux secteurs touchés de plein fouet par la crise de la covid-19. Je souhaite débuter mon intervention en saluant le travail remarquable mené par les structures associatives : sans elles, de très nombreux concitoyens se seraient retrouvés totalement démunis face à la crise et au confinement. Il me tient également à coeur de rendre hommage aux bénévoles de notre pays, qui n'ont pas compté leur temps pour apporter aide et soutien. Enfin, je tiens à saluer les jeunes, qui se sont fortement mobilisés pendant cette période, malgré les difficultés qui les touchent. Le ministre de l'éducation nationale indiquait samedi dernier, dans cet hémicycle, que la jeunesse devait être la « première de toutes les priorités ». Force est de constater qu'il est difficile d'en retrouver la traduction budgétaire dans ce programme 163. Bien évidemment, les crédits du plan de relance sont à saluer. Mais, à y regarder de plus près, plus de 80 % de l'effort pour la vie associative et la jeunesse est consacré au seul service civique et aux 100 000 missions supplémentaires annoncées. Le service civique est un très beau dispositif qui a fait ses preuves depuis sa création, en 2010. Toutefois, est-il réellement envisageable d'atteindre un objectif de 250 000 missions en une année, soit la moitié de ce qui a été réalisé en dix ans ? Le service civique ne saurait être, en ces temps de crise, une substitution à l'emploi. Il ne faudrait pas que le quantitatif prime sur la qualité des missions et de l'accompagnement. Par ailleurs, ces crédits ne sont que conjoncturels et n'ont pas vocation à aider durablement la jeunesse et le tissu associatif, qui en auraient pourtant fort besoin. Près de 30 000 associations seraient menacées de disparition en 2020. Concernant les crédits spécifiques du programme 163, la hausse de 6 % par rapport au budget pour 2020 s'explique quasi exclusivement par la montée en puissance du service national universel, le fameux SNU. C'est donc une augmentation des crédits en trompe-l'oeil, alors même que de fortes interrogations demeurent sur la mise en oeuvre, le déploiement et le fonctionnement du SNU. Son expérimentation n'a pas pu être menée à bien, la phase de cohésion n'a pu se tenir et le nombre de jeunes concernés reste particulièrement limité. limité. À cela s'ajoutent une mauvaise estimation du coût du SNU et une difficulté à percevoir sa coordination avec les autres politiques en faveur de l'engagement des jeunes. C'est pourtant un élément clé, au même titre que la formation des encadrants et l'implication du secteur associatif et des collectivités territoriales, peu associées jusqu'à présent. Pourtant, face à ce constat, à l'heure où notre pays traverse une crise majeure, alors même qu'il y a eu une sous-exécution des crédits de l'ordre de 20 millions d'euros cette année pour le SNU, le choix a été fait de doubler les crédits de cette action, avec l'inscription de 62,3 millions d'euros en 2021, soit 32,5 millions d'euros supplémentaires. Était-ce bien la priorité du moment ? Ces crédits auraient pu être affectés à des actions prioritaires au regard des urgences du secteur associatif, confronté à l'annulation de ses événements, à la baisse du nombre de cotisations, aux urgences du tourisme social, avec une activité quasi nulle des colonies de vacances, ou encore à l'urgence que représente la détresse de notre jeunesse. Voilà quelques jours, des présidents d'université évoquaient une « bombe à retardement sociale et humaine », en parlant de la situation des étudiants, confrontés à l'isolement, aux difficultés financières, à la perte de leur emploi et à une réelle détresse psychologique. En tant que sénatrice du Bas-Rhin, j'ai été marquée par ces files d'attente de jeunes, toujours plus nombreux, à Strasbourg, pour obtenir des produits de première nécessité. Je tiens à ce titre à saluer ici l'élan de solidarité et les actions engagées par les associations étudiantes, les artisans, les restaurateurs, les représentants professionnels, les collectivités territoriales et toutes les structures associatives qui se mobilisent en Alsace, comme partout en France, depuis des mois, pour leur venir en aide.

la priorité du moment, car nos jeunes ont besoin de retrouver des perspectives et des marques de confiance. La priorité, c'est aussi nos associations, dont nous savons à quel point elles contribuent à la solidarité, à la cohésion nationale et au lien social, si importants en ces temps compliqués.

nous vivons une crise sanitaire sans précédent, qui met à rude épreuve nos hôpitaux et notre personnel hospitalier, dont je tiens à saluer devant vous la remarquable implication. Cette crise sanitaire inédite nous affecte tous, altère notre capacité à vivre ensemble et à nous réunir. C'est pourquoi le rôle du sport, fondamental pour la santé et la cohésion sociale, résonne plus que jamais. J'ai entendu le cri des 360 000 associations sportives, qui ne peuvent pas jouer leur rôle dans cette période de confinement et craignent de devoir rembourser

Depuis samedi dernier, tous les adultes peuvent pratiquer de nouveau une activité sportive individuelle, dans la limite de trois heures et de vingt kilomètres autour de leur domicile. Ils peuvent accéder aux équipements de plein air.

crise économique majeure, à laquelle nous devons faire face. Tous les acteurs du sport étaient réunis la semaine dernière autour du Président de la République, qui a annoncé des mesures fortes pour le secteur sportif, au-delà des 3 milliards d'aides de droit commun débloqués depuis le début de la crise pour le sport amateur, le sport professionnel, le sport associatif et le secteur marchand. Nous avons mesuré l'urgence, pour le monde associatif et le monde du sport, et les difficultés qu'ils ont rencontrées depuis le mois de mars. Nous avons fait le nécessaire.

afin que nous arrivions progressivement à remplir des enceintes plus importantes dès que la situation sanitaire le permettra. Nous n'avons pas oublié les petites associations gérées par les bénévoles

Cette progression globale du budget, on le sait, s'inscrit dans un élan vers les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, qui représentent une véritable opportunité que nous devons saisir. Les 105 millions d'euros supplémentaires du programme 305 sont majoritairement alloués à la Solideo,

Je pense également aux très nombreux sites labellisés « centres de préparation aux Jeux », qui accueilleront les délégations avant les jeux Olympiques. Il s'agit aussi d'un héritage immatériel et durable pour notre pays et nos concitoyens.

Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs,

qu'une fraction de l'effort de la Nation, une fraction de tous les domaines dans lesquels l'État joue un rôle essentiel d'impulsion, d'innovation, de professionnalisation, de coordination et d'expertise. Avec un total s'élevant à 699,73 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, le programme 163 bénéficie, en dehors du plan de relance, d'une progression de ses ressources de près de 6 % par rapport à l'année dernière. Je souhaite vous présenter ce programme en trois points bien distincts, mais représentatifs de mon action en faveur de la jeunesse, de l'engagement et de la vie associative. Concernant la jeunesse, trois mesures méritent d'être mises en avant : l'accès des jeunes à l'information, qui bénéficie de 6 millions d'euros, la promotion des mobilités internationales, avec 17 millions d'euros pour l'OFAJ et l'OFQJ, et le développement des loisirs éducatifs de qualité pour la jeunesse, le soutien à l'éducation populaire, ou encore le tourisme social.

ici, en préambule, la grande mobilisation de notre jeunesse, qui a été saluée par un certain nombre de sénateurs et de sénatrices. Cette mobilisation a été à la hauteur de la crise. Notre jeunesse a été au rendez-vous, elle s'est mobilisée très largement

J'ai eu l'honneur de porter le transfert des Creps aux régions, mais avec les moyens adaptés. Cette mesure avait été adoptée par l'ensemble de la représentation nationale. J'ai le sentiment que M. Claude Évin n'aimerait pas ce budget, madame la ministre des sports : c'est de l'enfumage

immense pour toute une génération, dont la mienne. Le retour obligatoire aux casernes, pendant un mois, n'est pas satisfaisant. Les jeunes ne veulent pas apprendre à saluer d'une matière militaire ou rester au garde-à-vous. Ce qu'ils veulent, c'est se sentir utile, utile aux autres, à leur collectivité, à la Nation et à la planète. Le service civique remplit parfaitement ce rôle et doit être renforcé.

la rencontre de l'autre et, ainsi, la découverte de son altérité et de son humanité. C'est précisément pour cette raison que la mission Ruralité, à laquelle j'ai eu l'honneur de participer et qui avait vocation à

d'un Erasmus rural. Dans les territoires ruraux plus qu'ailleurs, les choix d'orientation des jeunes sont surdéterminés non seulement par des raisons financières, mais aussi par l'offre de formation locale, qui les conduit souvent à restreindre leurs ambitions. La création d'un Erasmus rural permettrait à des jeunes ruraux sans emploi ni formation de partir à l'étranger

qui sont, à la différence des biens matériels, les seules richesses que les civilisations produisent pour l'humanité tout entière. Tel est le sens de cet amendement gagé sur les crédits du SNU. Les deux amendements

Partout en France, nous avons vu plusieurs associations s'organiser, s'adapter, pour protéger leurs salariés et leurs bénévoles et poursuivre leurs activités lorsque cela était indispensable. Elles interviennent en relais de l'action de l'État

afin de venir en aide aux entités les plus en difficulté du fait de la crise sanitaire. L'augmentation de ce budget serait aussi un rattrapage des moyens perdus en matière de soutien aux associations à la suite de la suppression de la réserve parlementaire. Il s'agit donc d'augmenter de 50 millions d'euros les crédits consacrés au Fonds pour le développement de la vie associative afin d'aider les associations à faire face aux conséquences de la crise. Sans associations,

à l'été et à l'automne 2020 pour répondre à la déscolarisation d'un certain nombre d'enfants et qui s'est avéré très intéressant, permettant des avancées significatives- 125 000 enfants et jeunes ont été concernés. Valorisant notamment la découverte du patrimoine et l'éducation à l'environnement, les centres de loisirs et les colos apprenantes ont été sources de dynamisme pour leurs territoires d'implantation.

Alors que 4 millions d'enfants sont privés chaque année de vacances et que la crise économique et sociale que nous traversons s'aggrave, la pérennisation des actions en faveur des vacances et des loisirs éducatifs relève de l'utilité publique. Nous proposons donc le maintien de cette opération pour l'année à venir. libellé : La parole est à Mme Sabine Van Heghe Cet amendement vise à augmenter les moyens destinés au financement des clubs sportifs et des équipements dans les territoires qui sont fortement impactés par la crise sanitaire, une majoration de la subvention versée à l'Agence nationale du sport. Cette mesure est d'autant plus nécessaire qu'elle interviendrait confinement. Dans ce contexte sanitaire particulier, le retour au sport est un enjeu majeur pour la santé des jeunes et de tous les Français. M. Jean-Jacques Lozach. Le présent amendement vise à abonder les crédits du programme « Sport » à hauteur de 25 millions d'euros, afin de financer l'expérimentation d'un Pass'Sport. Cette expérimentation concernerait 50 000 jeunes volontaires. À la sortie de plusieurs mois de confinement et dans un contexte de crise sanitaire durable, la sédentarité chez les jeunes constitue un enjeu majeur de santé publique. En 2017, déjà, la Fédération française de cardiologie

Le Pass'Sport aurait pour objectifs de lutter contre le décrochage sportif et la sédentarité des jeunes, ainsi que de démocratiser la pratique sportive. Il serait accessible une application et ouvert ouvert aux 14-20 ans, soit la tranche d'âge couvrant les trois principales périodes de décrochage de la pratique sportive observées chez les jeunes, en particulier les jeunes filles : l'entrée en classe de quatrième, le passage du collège au lycée et le passage dans l'enseignement supérieur.

et bien communiquer, en tirant notamment les enseignements des difficultés rencontrées par le pass culture. En tout cas, si l'on attend un hypothétique PLFR, au mois de mai ou de juin 2021, pour financer le Pass'Sport,

de plein fouet par la crise sans précédent que traverse notre pays et sont confrontés à l'isolement, à la perte de repères, à la perte de perspectives et aussi à la précarité financière. L'impact psychologique du confinement doit également être pris en compte,

ou pour le paiement de leur loyer. Ils sont de plus en plus nombreux à se rendre au Secours populaire ou aux Restos du coeur, à frapper à la porte de structures associatives, pour y chercher de l'aide alimentaire, vestimentaire ou informatique. L'engagement des associations et des collectivités territoriales, ainsi que les initiatives qui ont émergé localement ont permis de pallier l'urgence, mais cela ne saurait suffire à faire face à cette situation particulièrement dramatique.

être utile, mais il a ses limites ... L'amendement n° II-700 a des qualités : il vise à abonder de 30 millions d'euros les crédits destinés au soutien au mouvement sportif : clubs, mais aussi équipements dans nos territoires. J'y suis favorable pour trois raisons.

En cas de non-versement ou de moindre versement des droits télévisés du championnat de France de football professionnel, c'est l'Agence nationale du sport qui en supportera toutes les conséquences. Il convient donc d'anticiper ce risque. Pour ce qui concerne tous les amendements

Une aide à la demande de sport sera ainsi distribuée aux familles, aux Françaises et aux Français, pour qu'ils retrouvent le chemin des clubs dès que la situation sanitaire permettra de refaire du sport normalement. Sachant que certaines personnes en difficulté ne pourront pas retourner dans des clubs,

d'abonder les crédits en faveur du sport pour tous. J'en profite- je ferai ainsi d'une pierre deux coups, monsieur le président -pour dire que nous avons rectifié notre amendement qui visait à abonder les crédits de la vie associative, de sorte que nous puissions en même temps

Vous avez le droit de défendre le SNU, chacun en pense ce qu'il veut, mais soyons honnêtes : le Président de la République lui-même, il y a deux jours, lorsqu'il a reçu le président du Sénat et les présidents de groupe,

nous préférons cibler les 30 millions d'euros du SNU sur des missions en direction de la jeunesse, des vacances apprenantes et des colonies de vacances. Nous espérons que les 100 millions d'euros que nous avons votés en première partie resteront bien affectés à l'Agence nationale du sport pour financer toutes les missions que vous avez citées, aussi bien au niveau des clubs qu'au niveau des fédérations.

proviennent du redéploiement de l'argent qui se trouve aujourd'hui encore dans les caisses de l'Agence nationale du sport. Vous imaginez bien que, en cette période où beaucoup d'événements ont été reportés, voire annulés,

du sport de nos territoires, auquel nous sommes particulièrement attachés. N'oublions pas non plus que l'environnement de cet écosystème est profondément touché. Je ne donnerai qu'un seul exemple, celui de l'UCPA, qui est le numéro un des loisirs sportifs en France et qui connaîtra une perte de 110 millions d'euros cette année.

par la fierté retrouvée et ainsi contribuer à l'estime de soi, qui est le moteur de l'émancipation individuelle et collective. C'est un amendement auquel je tiens. Je pense que l'on pourrait faire une expérimentation au moins au cours de l'année 2021. Je suis prêt à le modifier

et ainsi poser la première pierre de la mise en place d'une réelle politique publique d'insertion par le sport. Malheureusement fragilisées par la suppression des emplois aidés, les associations sportives oeuvrent au quotidien sur l'ensemble du territoire national en accompagnant les jeunes en difficulté. Elles participent à la mixité sociale et créent du lien dans des territoires difficiles. Elles apportent des réponses concrètes aux attentes des jeunes.

Ce serait une solution pertinente pour sensibiliser la jeunesse à la culture et aux traditions françaises, en répondant aux enjeux de résilience et de sécurité alimentaire actuels, à la dégradation de la biodiversité et aux besoins d'adaptation aux dérèglements climatiques. L'objet de cet amendement est de revaloriser le secteur agricole, promouvoir l'agroécologie, de sensibiliser les Français dès leur plus jeune âge à l'alimentation durable, ainsi qu'aux enjeux liés à la préservation de l'environnement, de la diversité biologique

Van Heghe. Cet amendement vise à redéployer des moyens en les fléchant en direction du soutien à la vie associative sportive dans les QPV et dans les zones de revitalisation rurale. Il s'agit ainsi de promouvoir un certain nombre d'actions en faveur de l'éducation et de l'insertion Nous proposons de concentrer nos moyens dans les territoires où l'offre de pratique sportive est limitée. Par ailleurs, les populations les plus éloignées du sport- les publics socialement défavorisés, les jeunes, les publics féminins, les personnes en situation de handicap -représentent aussi un fort potentiel de développement du sport.

Stade de France. J'ai souligné les fragilités de la relation contractuelle entre l'État et le consortium du Stade de France dans un rapport publié en 2019. Pour autant, nous sommes tenus par nos obligations contractuelles. C'est pourquoi je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j'y serai défavorable.

Le secrétaire d'État chargé de la ruralité a annoncé la création de 800 postes de « volontaires territoriaux » pour soutenir les communes rurales dans leurs besoins en ingénierie. Afin de donner une impulsion aux projets mis en oeuvre dans le monde rural, il serait intéressant d'affecter des volontaires du service civique auprès de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Il s'agirait ainsi d'accompagner rapidement la mise en place de projets structurants permettant de conforter des économies locales, qui, comme on le sait, ont été très affectées par les conséquences de la pandémie. En outre, le développement d'un engagement citoyen auprès du monde rural pourrait susciter des vocations au sein de la jeunesse. Tel est l'objet de cet amendement, déposé par mon collègue Jean-Yves Roux. Quel est l'avis de la commission

Les crédits dédiés au service civique sont suffisants pour soutenir ce genre de dispositif. Le problème risque davantage de résider dans leur consommation effective, en particulier s'agissant des crédits ouverts au titre du plan de relance. L'avis est donc défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ?

la solidarité, la fraternité et la générosité. C'est aussi l'un des derniers havres de mixité sociale. Or ce monde est en danger, cela a été dit à de multiples reprises.

de loi de finances pour 2020. Les informations souhaitées sont essentielles pour apprécier et évaluer l'efficacité du dispositif mis en place dans la durée, et pas uniquement de façon ponctuelle. C'est pourquoi, pour ne pas avoir à adopter chaque année un rapport dédié, le présent amendement vise à compléter le contenu de l'annexe budgétaire relative à l'effort financier de l'État en faveur des associations, remise avec le projet de loi de finances de chaque année.

En cela, il ne saurait être rattaché à « l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques », seul fondement prévu par l'article 34 de la loi organique relative aux lois de finances du 1août 2001 pour une demande de rapport introduite en loi de finances. C'est pourquoi il est proposé de supprimer ce cavalier budgétaire.

ces travaux comportent des propositions ambitieuses visant à lutter contre la radicalisation dans le milieu sportif. Il n'est plus temps d'évaluer « la possibilité de renforcer les dispositifs existants et l'opportunité de créer de nouvelles mesures ». Il est temps d'agir Ce sera notamment l'objet du projet de loi confortant les principes républicains. Attendre encore un an est aujourd'hui inconcevable. C'est dans le cadre de ce texte à venir que de nouvelles mesures doivent être prises. Si le Gouvernement veut présenter sa politique et ses possibles évolutions, il est nécessaire que cela soit fait en amont de l'examen du projet de loi

cette politique correspondrait à une dépense annuelle de presque 2 milliards d'euros. Le présent amendement vise à demander au Gouvernement de présenter un rapport précis sur le SNU,

J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.